Je vous rappelle que, dans ce débat, le Gouvernement aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes ; l’orateur disposera alors à son tour du droit de répartie, pour une minute.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous le savons, la sécurité est une préoccupation majeure pour nos concitoyens. À l’heure où les guerres menacent aux portes de l’Europe, où nos quartiers et nos campagnes sont sous l’emprise des narcotrafiquants, où nombre de nos concitoyens rencontrent des difficultés pour se soigner, les sujets liés à notre sécurité individuelle ou collective saturent le débat public, qu’il s’agisse de la défense nationale, de la sécurité publique ou encore de la sécurité sociale. En dehors des grandes catastrophes naturelles ou accidentelles, la sécurité civile est moins souvent évoquée. Il existe pourtant en France un service public tout à fait exceptionnel pour garantir la protection de nos concitoyens et leur porter secours et assistance.

jusqu’à plusieurs centaines de femmes et d’hommes formés à toutes les spécialités de secours et équipés de moyens considérables, partout sur le territoire, à la ville comme à la campagne,

enfin, par son mode de financement, puisque les Sdis sont largement alimentés par les collectivités et, en premier lieu, par le département. Grâce à ce modèle, les Sdis assurent quotidiennement leurs missions de secours de proximité à travers un maillage territorial de 6 000 centres d’incendie et de secours, réalisant près de 5 millions d’interventions par an. Il s’agit d’un service public essentiel du quotidien, au cœur des valeurs républicaines de fraternité, de solidarité et d’engagement.

qui effectuent 67 % du temps d’intervention et ne représentent que 12 % des dépenses. C’est donc l’engagement citoyen qui constitue le socle du modèle français. Cette spécificité est aujourd’hui remise en cause par l’application de la directive européenne de 2003 sur le temps de travail, dont l’interprétation pour les sapeurs pompiers a été revue à la suite de la jurisprudence en 2018. Une requalification du statut des sapeurs pompiers volontaires, intégrant une obligation de professionnalisation, diminuerait considérablement le service rendu à la population. Nous pouvons sans peine anticiper les effets d’une telle évolution, notamment en milieu rural, de l’allongement du temps d’intervention ou bien encore de la forte augmentation du coût de la sécurité civile dans les finances publiques. S’il faut absolument conserver l’hybridité des statuts, il paraît en revanche

est caractérisée par une sursollicitation dans le domaine médical, au travers du volet « secours et soins d’urgence aux personnes ». Sur les 75 600 interventions menées en 2023 dans le département de la Loire Atlantique, les trois quarts relèvent de cette catégorie. Cette sursollicitation sur le secours à la personne met en exergue la fragilisation d’autres services publics de santé, la désertification médicale, la disparition de services hospitaliers d’urgence en milieu rural et les carences ambulancières, notamment.

Cette perte de sens se traduit aujourd’hui par une moindre attractivité de la profession, alors même que notre modèle de sécurité civile sera mis à l’épreuve, dans les années à venir, par l’augmentation des phénomènes climatiques critiques et par les évolutions démographiques.

particulièrement concernés par des problématiques climatiques spécifiques et lourdes. Face à ces risques d’ampleur croissante, l’ambition doit rester la même qu’aujourd’hui : il faudra conserver des capacités d’anticipation qui préservent en amont et des capacités d’adaptation qui sauvent pendant la crise. Cet objectif ne pourra être atteint que par une nécessaire consolidation du financement des Sdis.

Les principaux contributeurs sont les départements, qui assument la plus grande partie de la hausse des dépenses depuis 2003. Or leur situation budgétaire est extrêmement préoccupante, voire

Les communes, quant à elles, ne peuvent prendre le relais du fait du plafonnement de leur contribution. Les collectivités territoriales semblent donc avoir de plus en plus de difficultés à suivre la dynamique de dépenses des Sdis, dont les budgets sont principalement affectés aux ressources humaines. Dès lors, toutes les pistes doivent être explorées.

lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024 – ou encore par l’actualisation de son assiette, inchangée depuis 2003. La création d’une nouvelle part départementale, additionnelle à la taxe de séjour, qui associerait plus étroitement les touristes et les visiteurs au financement des services d’incendie et de secours mérite également d’être étudiée. Enfin, les travaux autour de la « valeur du sauvé » doivent être poursuivis. Car, dans les débats sur le modèle de financement des Sdis, la participation des assureurs, qui retirent un certain bénéfice des interventions menées, ne doit pas être oubliée.

sept ans. Pendant toutes ces années, j’ai vu des hommes et des femmes affronter tous les risques et faire preuve d’un courage et d’un dévouement remarquables, au détriment de leur vie professionnelle et familiale, et, parfois, hélas ! au péril

Ces événements, souvent imprévisibles, exigent une réponse rapide, efficace et adaptée. Face à cette multiplication des risques, il est crucial que nous soutenions nos services départementaux d’incendie et de secours, véritables piliers de la sécurité civile.

de toute l’Europe. Ces incendies, qui se déclarent plus tôt dans l’année et qui sont plus violents, représentent une menace de plus en plus grande pour nos territoires et pour nos forces de secours. Un point essentiel ne doit pas être oublié : la santé des sapeurs pompiers. En effet, plusieurs études ont révélé une réalité alarmante.

Ce dispositif fondé sur les contributions des départements et du bloc communal, exsangues financièrement, n’est plus tenable. Il y a urgence à inscrire dans la durée le soutien financier de l’État, en pérennisant notamment les pactes capacitaires des Sdis, à hauteur des engagements pris par l’État au lendemain des importants feux de 2022. Cela a été fait pour les

permettrait de se rendre compte de l’importance du travail réalisé et de la valeur des vies, de l’environnement et des biens sauvés. Mes chers collègues, il est urgent de mettre en place des solutions concrètes pour renforcer les capacités de nos Sdis. Le financement pérenne de ces services est un impératif absolu pour faire face aux risques actuels et à ceux qui viendront.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme un certain nombre d’entre nous dans cet hémicycle, j’ai eu la chance d’exercer la responsabilité de président de Sdis, de rencontrer des gens dévoués

Une épée de Damoclès pèse sur le statut du volontariat à la française. Depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne et l’avis rendu par le Comité européen des droits sociaux de février 2024, plane le risque que le sapeur pompier volontaire soit requalifié en travailleur.

(Samu) a pris la mauvaise habitude d’appeler ceux qui décrochent le plus vite et qui coûtent le moins cher, c’est à dire les pompiers. Ceux ci assument maintenant une bonne partie des transports sanitaires.

départementaux et municipaux, qui sont les contributeurs.

département très touristique, il me paraît important que des collectivités qui doublent ou triplent leur population à certaines périodes de l’année puissent augmenter leur taxe de séjour et en attribuer une part aux Sdis concernés.

Comment soutenir les Sdis dans leur gestion des nouveaux risques, au regard du financement de leurs missions ?

est de réduire les coûts d’achat de véhicules et de matériels pour les Sdis, de permettre l’émergence d’une offre française et européenne susceptible de répondre aux besoins de la lutte aérienne contre le feu, ainsi que de limiter la dépendance à l’égard d’un nombre restreint d’acteurs extérieurs. le groupe de travail a proposé de constituer une cellule « fonds européens » au sein de la DGSCGC. Elle disposerait de moyens humains dotés des expertises juridiques nécessaires pour servir de guichet unique national, destiné à faciliter l’accès aux fonds européens susceptibles d’être sollicités par les acteurs publics de la sécurité civile. En effet, en France, En effet, en France, le recours effectif aux financements européens demeure relativement limité dans ce domaine, contrairement à nos voisins. L’accès à ces subventions est souvent rendu difficile par la complexité des procédures

monsieur le ministre

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’actualité nous rappelle, une fois encore, combien les risques naturels et les menaces modernes nécessitent de notre part une vigilance accrue et des moyens renforcés. Les inondations récentes en Espagne, au bilan dramatique, mais aussi celles qui se sont déroulées en octobre dernier témoignent de la fréquence croissante de ces événements climatiques extrêmes. Je n’oublie pas, bien sûr, la multiplication et l’intensification des feux de forêt, qui inquiètent par leur ampleur et par leur caractère dévastateur. Surtout, ils ils surgissent désormais en des lieux et en des moments inattendus. Ces phénomènes, conséquence directe du bouleversement climatique, mobilisent nos services départementaux d’incendie et de secours bien au delà des périodes des amplitudes de risque ordinaires. Ils nous rappellent, certes, combien il est urgent de lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi de soutenir ces services essentiels à la sécurité des Français, d’autant que les catastrophes naturelles ne sont qu’une partie des défis actuels auxquels ces services doivent faire face. Les nouvelles menaces, qu’elles soient terroristes ou qu’elles impliquent des risques d’attaques chimiques et biologiques, exigent également une préparation et des moyens techniques et humains spécifiques. Dans ce contexte, les sapeurs pompiers sont appelés à être des acteurs de plus en plus polyvalents, capables d’intervenir dans des situations de crise variées et parfois inédites. À ce stade, je tiens à rendre hommage à nos 240 000 sapeurs pompiers, dont 80 % sont des dont 80 % sont des volontaires. Ils assurent, bien souvent au péril de leur vie, une mission essentielle. Aussi ai je une pensée émue pour celles et pour ceux qui, dans l’accomplissement de leur mission, ont perdu la vie ou ont été blessés. Face aux bouleversements évoqués, la mission des Sdis se transforme, pour répondre à la complexité croissante des interventions et à la diversité des risques. Cette adaptation nécessaire pèse immanquablement sur leurs dépenses, alors que ces services constituent déjà l’un des postes les plus dynamiques de la dépense publique. En effet, la modernisation des équipements, l’amélioration des conditions de travail et les revalorisations salariales, indispensables pour valoriser un engagement qui ne faiblit jamais, représentent des investissements coûteux. À l’heure actuelle, ce sont principalement les départements qui supportent cette charge. L’État assure environ un quart des financements des tandis que la participation du bloc communal s’est en partie déplacée vers l’intercommunalité. C’est dans ce contexte que nous débattons aujourd’hui du financement de la sécurité et du soutien à apporter aux Sdis dans leur gestion des nouveaux risques. Des évolutions notables ont été réalisées. Face à la recrudescence des feux de forêt, le Président de la République a pris l’initiative de renforcer la flotte aérienne, essentielle pour les interventions rapides. Face aux menaces modernes, de nouveaux équipements la formation des sapeurs pompiers et pour le développement de la coopération interservices, qui sont essentiels dans la gestion de crise. Notre assemblée a également été particulièrement active dans le soutien apporté aux Sdis dans l’exercice de leurs missions. Rappelons que l’exonération de taxe sur les carburants

budgétaire demeure élevée et la hausse des dépenses s’annonce difficilement tenable sur le long terme. Dans ce contexte, il est impératif d’explorer de nouvelles pistes pour réformer et soutenir le financement des car les collectivités semblent avoir de plus en plus de difficultés à suivre la dynamique de leurs dépenses. Les départements, principaux contributeurs au financement des Sdis, ne disposent que de faibles marges de manœuvre. Aussi faut il réfléchir aux moyens d’accroître les ressources financières

de pérenniser ce modèle auquel nos concitoyens sont profondément attachés. Je souhaite ici évoquer les centres de première intervention non intégrés plus particulièrement l’engagement de leur plus de 9 000 sapeurs pompiers volontaires. L’efficacité de notre modèle de sécurité civile repose en grande partie sur cet engagement, et il convient de leur témoigner notre reconnaissance. Pour soutenir cet effort, il conviendrait de sécuriser juridiquement la pratique de certains Sdis ou départements qui prennent en charge l’allocation de vétérance. Ouvrir plus largement cette possibilité permettrait de soulager les communes et, en même temps, de soutenir le volontariat. Mes chers collègues, face à tous ces défis, nous devons faire les choix stratégiques qui assureront aux Sdis les moyens d’assumer leur mission dans un contexte de risques croissants et complexes. La France dispose d’une sécurité civile qui est d’un haut niveau d’excellence, mais cet atout dépend de notre engagement à pérenniser et à renforcer ce modèle. Plus que jamais, nous devons engager les réformes nécessaires au soutien et à la valorisation de ces services indispensables à notre sécurité. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà à quelques jours d’une relance du Beauvau de la sécurité civile, prévue le 25 novembre prochain. J’y vois, monsieur le ministre, l’occasion de vous faire part des préoccupations les plus concrètes des territoires ruraux.

repose à 96 % sur l’engagement de sapeurs pompiers volontaires. L’épée de Damoclès d’une possible requalification du statut fait craindre le risque d’un effondrement. Nous devons lever ces incertitudes le plus rapidement possible. Mes chers collègues, nos Sdis sont arrivés à un point de rupture, et ce d’autant que les collectivités locales, départements en tête, contributrices à hauteur de 5,6 milliards d’euros, sont exsangues. Or la sécurité civile ne saurait être une variable d’ajustement budgétaire

signifie 230 000 euros de recettes en moins. Le bilan est simple : un endettement accru et l’impossibilité de renouveler le matériel. Est ce bien prudent ? Est ce juste ? juste ? Ce n’est pas nouveau, mais cela devient urgent : des mesures structurelles de bon sens s’imposent, au premier rang desquelles la mutualisation et – son corollaire – la péréquation. Deuxième piste d’action : la rationalisation de la commande publique et une exigeante simplification administrative et normative.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les récentes inondations qui ont ravagé l’Espagne et nombre de départements français rappellent, s’il en était encore besoin, le caractère vital des services d’intervention en cas de catastrophe naturelle. Dans notre pays, ce sont les services départementaux d’incendie et de secours qui sont au centre du dispositif d’aide aux victimes. Leur excellence n’est plus à prouver, comme en témoigne la position de la France comme premier contributeur du mécanisme de protection civile de l’Union européenne. Aujourd’hui, les Sdis sont cependant menacés par un effet de ciseau. D’un côté, les besoins ne vont malheureusement pas cesser d’augmenter. Le changement climatique, en particulier, ne peut que multiplier l’occurrence et l’intensité des phénomènes climatiques extrêmes, qu’il s’agisse des tempêtes ou des feux hors norme. On peut également penser au phénomène de retrait gonflement des argiles, qui va fragiliser un nombre considérable de bâtiments sur le territoire national ; et je n’oublie pas la lutte contre les risques industriels et technologiques. D’un autre côté, dans le contexte budgétaire que l’on connaît, les moyens financiers qui sont alloués aux Sdis tendent à stagner, voire à régresser.

Pour intéressantes que soient ces pistes côté dépenses, elles ne régleront pas structurellement le problème : nous ne pouvons faire l’économie d’une réforme du financement des Sdis. Je remercie donc nos collègues du RDSE d’avoir inscrit cet indispensable débat à l’ordre du jour de la Haute Assemblée.

plusieurs leviers peuvent être actionnés pour en augmenter le rendement. Deuxièmement, on peut envisager le versement aux Sdis d’une quote part de la taxe de séjour et la création d’une contribution nouvelle sur les locations de type Airbnb.

élargissement serait délicat pour les collectivités, alors même que, en la matière, la solidarité nationale devrait jouer à plein. C’est pourquoi la quatrième piste me semble plus intéressante. Elle recouvre deux voies plus originales qui pourraient être explorées :, l’élargissement de la possibilité de facturation par les Sdis de prestations qui

dernières pistes sont véritablement disruptives, car elles impliquent en quelque sorte un changement de culture de la part des Sdis. Mais, face à la montée en puissance des périls naturels, il va falloir se résoudre à décloisonner le secteur public et le secteur privé en matière d’intervention et de secours.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, parmi les nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les services départementaux d’incendie et de secours, que l’ensemble de nos sapeurs pompiers, qu’ils soient professionnels ou volontaires, on pense évidemment aux effets du changement climatique. Celui ci s’accélère. L’observatoire européen Copernicus vient de le démontrer 2024 sera la plus chaude jamais enregistrée. Dans tous nos départements, nous connaissons désormais trop bien les conséquences d’un tel état de fait : inondations, feux de forêt, crues, tornades, canicule, sécheresse…

le Sdis de Seine Maritime a dû réaliser près de 600 interventions pour les seules journées des 2 et 3 novembre. Les conséquences du dérèglement climatique poussent également les Sdis à adapter leurs techniques et à renforcer leurs moyens et ressources. En plus de développer la formation, ils doivent désormais se doter de nouveaux équipements nécessaires à la lutte contre des risques auxquels ils étaient autrefois peu confrontés. Ces évolutions devraient accroître les coûts qu’ils supportent Parmi les nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les sapeurs pompiers, il y a aussi la désertification médicale et les difficultés de nos services de santé à assumer leurs missions – je pense en particulier aux carences ambulancières. Lorsque les services d’urgence ferment régulièrement,

communes et intercommunalités pourront répondre aux besoins des Sdis, en fonctionnement, en équipement, en matériel, en véhicules, etc. d’autant que, en parallèle, ce même projet de loi de finances affiche une baisse

comment les départements pourront ils encore financer et soutenir les Sdis dans leur gestion des nouveaux défis et des nouveaux risques ? Face à l’augmentation de la population et à l’émergence de risques liés au dérèglement climatique ou à l’évolution de la menace, il apparaît aujourd’hui indispensable de réformer le mode actuel de financement

Ce rapport met en lumière la polyexposition de nos pompiers à des substances toxiques, dont certaines sont reconnues comme cancérogènes, telles que les fumées toxiques, l’amiante, les retardateurs de flamme, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), les perturbateurs endocriniens, les protoxiques ou les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Pour répondre au développement de ces risques, le rapport préconise d’élargir la présomption d’imputabilité au service aux types de cancer dont le lien avec l’activité de sapeur pompier est reconnu par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ), comme le font d’autres pays tels que le Canada, les États Unis ou encore l’Australie.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la sécurité civile, fondement de notre République, repose sur une organisation à même de répondre efficacement aux besoins spécifiques de nos territoires.

Beaucoup de territoires ultramarins font face à tous ces défis. Les risques naturels, notamment les cyclones et les inondations, combinés aux exigences liées à l’activité portuaire et touristique, appellent une organisation locale plus réactive et adaptée.

du seul centre de secours de l’île implique une autosuffisance opérationnelle en cas de catastrophe majeure, dans l’attente des premiers renforts.

puisque nous disposerons de notre propre schéma territorial d’analyse et de couverture des risques (Stacr). Avec une administration autonome et un niveau opérationnel en phase avec les enjeux, à même d’anticiper une gestion opérationnelle sans faille en attendant l’arrivée des renforts et de répondre à la crise du volontariat, qui touche tous les territoires français.

ces dernières, surtout les ultramarines, font face à des contraintes budgétaires importantes, amplifiées par l’insularité. Ainsi, le coût de fonctionnement de notre Stis est estimé à plus de 9 millions d’euros, charge qui incombera

Celles ci cumulent les compétences d’une commune, d’un département et d’une région, mais avec des ressources financières limitées par leur statut. Cette spécificité renforce la nécessité d’un accompagnement de l’État, car il est primordial que la collectivité puisse assumer cette responsabilité sans compromettre la réalisation d’autres priorités essentielles pour le territoire. Les besoins sont clairs et nombreux : renouveler les équipements obsolètes, recruter du personnel administratif pour répondre à la création des différents services, renforcer la formation des sapeurs pompiers, proposer des mesures incitatives pour fidéliser les sapeurs pompiers volontaires

et adaptée face aux risques, requiert donc le soutien financier de l’État. La sécurité civile est un droit fondamental, dont la réussite repose sur des choix clairs et ambitieux. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les débats sur le financement de nos politiques publiques ont pris une acuité toute particulière ces derniers mois. C’est dans ce contexte, que chacun a bien à l’esprit,

contexte financier est difficile. J’ai essayé, en préparant mon intervention, de rester fidèle à ma ligne, c’est à dire de ne pas proposer de prélèvement obligatoire supplémentaire.

De manière plus structurelle, l’augmentation de la demande opérationnelle dans le domaine sanitaire progresse bien plus vite et plus fortement que les ressources. Forcément, cela coince… Le vieillissement de la population et les déserts médicaux grandissants viendront encore renforcer cette pression opérationnelle sur le secours aux personnes. En ce qui concerne les recettes, les premiers financeurs des Sdis que sont les départements sont eux mêmes asphyxiés.

Que ce soit en raison des menaces pesant sur l’engagement non professionnel ou de l’application de la directive européenne sur le temps de travail, l’affaissement du volontariat imposerait de recruter immédiatement des sapeurs pompiers professionnels, dont nous ne saurions pas aujourd’hui financer les postes. Voilà, à mon sens, le premier risque auquel s’attaquer pour éviter la remise en cause non seulement de notre modèle de sécurité civile, mais aussi de son financement. financement. Les nouveaux risques de sécurité civile, à proprement parler, ont déjà été analysés : extension dans le temps et dans l’espace des feux de forêt et d’espaces naturels, inondations, risques liés à la protection de notre patrimoine ou au développement des motorisations électriques.

La parole est à Mme Nadine Bellurot, pour le groupe Les Républicains.

sans nos sapeurs pompiers professionnels et, tout particulièrement, volontaires, nous ne pourrions pas faire face aux conséquences de la désertification médicale. Ils comblent en grande partie les défaillances du système de santé, alors que l’Indre fait partie des territoires les moins bien dotés. Pour leur engagement sans faille, je souhaite donc les saluer et les remercier. Tous les Sdis sont confrontés à un accroissement du nombre de leurs interventions, notamment au titre du secours d’urgence aux personnes, soit environ sept interventions par minute. Comme

En parallèle, les Sdis doivent s’adapter aux nouveaux risques et aléas liés au changement climatique. En témoigne, ces dernières années, l’accroissement des feux d’espaces naturels résultant des fortes chaleurs et des sécheresses. En 2021, dans le parc naturel régional de la Brenne, dans le département de l’Indre, près de 100 hectares ont été détruits par les flammes, alors que ce département, historiquement, n’est pas un territoire en proie aux incendies.

aux sapeurs pompiers. Ces derniers appellent d’ailleurs à une meilleure préparation des territoires pour faire face à ces risques aujourd’hui étendus. Ainsi, de nombreux Sdis évoquent

par l’action préventive des sapeurs pompiers. On peut citer le bâchage en période d’inondation ou encore la préservation des massifs forestiers et des milliers d’hectares épargnés des flammes grâce aux moyens des Sdis.

de couverture. Cela a permis non seulement de sécuriser les logements et infrastructures menacés à la suite des intempéries, mais également d’éviter des dégâts supplémentaires. Par voie de conséquence, l’intervention du Sdis, en se substituant à celle d’entreprises privées, réduit les coûts des compagnies d’assurances qui y auraient fait appel. Dans Dans le contexte budgétaire que vous connaissez, il est demandé aux collectivités territoriales de participer à l’effort de redressement des comptes publics. Rappelons pourtant que les premiers financeurs des Sdis sont les conseils départementaux, les communes et les intercommunalités.

avec les compagnies d’assurances en vue de reverser aux Sdis une part de cette portion « sauvée » ? Cela permettrait de les rétribuer à hauteur d’une partie du coût réel des dégâts ou dommages

de notre chaîne de sécurité depuis 1996. Je veux saluer l’intelligence des territoires : les présidents de conseils départementaux, les présidents des conseils d’administration des Sdis, les maires et les préfets ont su inventer un modèle de gouvernance robuste, réactif et résilient. Les résultats sont au rendez vous. En témoigne la capacité de mobilisation des sapeurs pompiers, qui interviennent

notre modèle a un coût et nous savons qu’il va falloir trouver de nouvelles sources de financement, en lien avec les principaux financeurs que sont les départements, les communes et l’État. Le budget national des Sdis, d’un montant de 6 milliards d’euros, est financé à près de 60 % par les conseils départementaux,

Pour pérenniser ce modèle unique au monde, nous devons valoriser l’engagement des sapeurs pompiers volontaires et avoir des gestes forts de reconnaissance de leur action au service de la Nation.

évidemment, nous y associerons les associations agréées de sécurité civile, également concernées par les questions de valorisation et de reconnaissance de leur engagement bénévole,

Le ministre de l’intérieur s’est engagé hier, devant la commission des lois du Sénat, à tenir les engagements pris pour renouveler la flotte d’hélicoptères EC145. La question des avions bombardiers d’eau se pose également. Il est de notre responsabilité collective de trouver des solutions soutenables financièrement pour garantir à la fois notre résilience et notre souveraineté. Préserver notre modèle de sécurité civile, sécuriser le financement des Sdis et se préparer au dérèglement climatique sont les défis que nous devons relever ensemble. Dans cette perspective, vous pouvez compter sur le Gouvernement et sur moi

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

les événements d’ampleur extraordinaire sont de plus en plus fréquents, en particulier les phénomènes de crues soudaines. Les inondations dramatiques que nous avons connues ces dernières années,